qui a remplacé Philippe Tabarot, nommé ministre. Au nom du Sénat, je lui souhaite la bienvenue parmi nous. Je salue également le retour de nos collègues Agnès Canayer et Laurence Garnier, que nous sommes

Il avait 14 ans, il rentrait d’un entraînement de foot. Il n’aura jamais 15 ans, parce qu’il a trouvé sur sa route deux adolescents délinquants récidivistes qui en voulaient à son téléphone portable et l’ont poignardé. J’ai, bien sûr, une pensée pour sa famille et pour ses proches. Ces deux délinquants étaient connus de la justice des mineurs, l’un pour des vols avec violence et port d’arme blanche, l’autre pour violence en réunion. Pour ces faits, ils avaient été présentés à un juge le 30 octobre 2024, en vue d’un jugement définitif prévu pour juin 2025.

ceux qui sont responsables de cette situation, les jeunes mineurs violents, mais également de comprendre ce qui ne va pas dans notre justice des mineurs – vous avez parfaitement raison. Ce qui ne va pas, monsieur le sénateur, se résume

Pendant que le CAC 40 reverse 100 milliards d’euros à ses actionnaires, les plans de licenciement s’accumulent dans toute la France, y compris dans des entreprises rentables. Michelin, la Fonderie de Bretagne, General Electric, ArcelorMittal, Photowatt : au total, la CGT a recensé 300 plans en cours, soit un total de 300 000 emplois menacés. Alors que le chômage a augmenté de 3,9 % au dernier trimestre, une hausse inédite en dix ans, votre doctrine reste inflexible : poursuivre le libre échange et la politique de l’offre, c’est à dire distribuer des milliards sans aucune stratégie ni contrepartie !

les salariés et les élus locaux, de manière transpartisane, réclament une nationalisation temporaire pour relancer l’activité. Le coût d’une telle mesure a été chiffré à 200 millions d’euros. En comparaison, l’utilisation de sel importé implique des essais de validation de missiles nucléaires dépasse le milliard d’euros ! Et je ne parle pas de la dépollution des sites industriels et des risques environnementaux liés au transport de matières dangereuses… Monsieur le ministre, ne pas agir, c’est faillir ! Avec la nationalisation, vous avez entre les mains un outil unique de planification.

pour évoquer, avec les élus locaux et les représentants des salariés, ce dossier révélateur des difficultés que traverse notre industrie. Je veux d’abord dire combien nous sommes mobilisés pour garantir notre souveraineté industrielle.

La parole est à Mme Marie Claire Carrère Gée, pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, mes chers collègues, si Élias est mort, c’est notre faute à tous. Je suis la mère de deux enfants, qui ont chacun leur tour été rackettés, violemment, dans le XIV arrondissement de Paris. J’ai essayé de les convaincre de ne jamais jouer les héros face à des racketteurs. Je n’en ai pas honte : je voulais juste être sûre qu’ils rentrent à la maison. Mais je veux me battre, parce que telle n’est pas du tout la société dans laquelle j’ai envie de vivre.

Deuxièmement, la punition va de pair avec l’éducation. Actuellement, on ne marche que sur une jambe ! La loi interdit de fait les courtes peines de prison. Il n’existe que six centres pénitentiaires pour mineurs et cinquante quatre centres éducatifs fermés, qui ne sont d’ailleurs

on n’y pense même plus ! Quatrièmement, l’excuse de minorité devrait être motivée par le juge pour chaque affaire. Bien sûr, les mineurs ne sauraient être par principe jugés comme des adultes – cela va de soi. Mais ils ne sauraient non plus être

Aujourd’hui, madame la ministre, le gouvernement dont vous faites partie a annoncé revenir sur ces transferts de charge. Pourtant, la hausse du prix des complémentaires demeure quant à elle bien réelle pour nos concitoyens. Dans notre rapport, nous avions formulé plusieurs propositions concrètes.

La parole est à M. Daniel Chasseing, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. Monsieur le président, monsieur le ministre de la souveraineté industrielle, mes chers collègues, l’hydroélectricité couvre 25 % des besoins de la France lors des pics de consommation. Elle est

la matière a un impact sur le fonctionnement électrique, qui souffre d’un manque de capacité de stockage. Le nombre d’heures vendues à prix négatif a été multiplié par trois en 2024. Nous devons donc lancer de nouveaux projets de Step. Mais, pour ce faire, il faut sortir de la concession.

européens. Il permettrait de sortir du blocage de la Commission européenne, qui dure depuis longtemps, et de relancer l’investissement dans les Step. Monsieur le ministre, pourquoi un tel retard ? Le régime de l’autorisation est en vigueur dans de nombreux pays !

Vous avez mentionné les solutions qui sont à l’étude : modifier la directive Concessions de 2014, mettre en place une régie ou une quasi régie ou encore basculer vers un régime d’autorisation.

Or, plus que par le passé, sans aucun doute, ce budget en détermine 35 000 autres : celui de nos collectivités locales, mairies et intercommunalités, qui attendent de savoir sur quelles bases elles pourront fonder leurs actions de proximité, mener à bien des investissements et soutenir une économie qui vacille.

qui se sont tenues au Sénat le 9 octobre dernier, l’ancien Premier ministre Michel Barnier indiquait vouloir mettre un terme au transfert obligatoire de ces deux compétences aux intercommunalités en 2026, sous réserve que les transferts n’aient pas encore été réalisés. Quant au Premier ministre François Bayrou, il a déclaré le 14 janvier dernier : « Mon gouvernement confortera les avancées sur des sujets très attendus comme l’eau [et] l’assainissement. » Or, mes chers collègues, le 1 janvier 2026, c’est demain demain, les exécutifs locaux devront effectuer des études ou y renoncer, décider, apprécier le prix de l’eau, les périmètres d’action, délibérer, recruter, prévoir des budgets en conséquence, ou au contraire ne pas les prévoir.

La différenciation territoriale est d’ailleurs l’un des principes du plan Eau qui avait été présenté par le Président de la République en septembre 2023. Rien à voir ! C’est pourquoi je suis favorable, pour les collectivités locales qui n’y auraient pas déjà procédé, à la suppression de l’obligation de transfert vers les EPCI des compétences eau et assainissement.

messieurs les ministres, mes chers collègues, je ne peux rester silencieux après les propos tenus par le Premier ministre lundi soir et réaffirmés hier devant l’Assemblée nationale, en réponse à Boris Vallaud., propos copieusement applaudis par les députés du Rassemblement national, le regard gourmand et le sourire aux lèvres ! Je ne peux me résoudre à ce qu’un Premier ministre qui doit tout au front républicain se laisse submerger par le vocabulaire de l’extrême droite. Les étrangers représentent un habitant sur dix dans notre pays. Ne vous laissez pas submerger par les fantasmes et les contrevérités ! Non, la France n’est pas submergée par l’immigration. Le rôle d’un Premier ministre n’est pas d’attiser les peurs, c’est de dire la vérité aux Français. Cette question doit être abordée dans un climat apaisé, sans tomber ni dans l’angélisme ni dans l’amalgame. Ce n’est pas un tabou ! Socialistes, nous regardons la réalité en face. Oui, l’immigration doit être inclusive et raisonnée. Oui, il manque aujourd’hui de véritables politiques d’intégration. Il faut traiter cette question sérieusement, et non en stigmatisant celles et ceux qui ont fait le choix, souvent contraint, de s’installer sur notre sol, d’y fonder leur famille et d’y construire une nouvelle vie. eux, qu’en serait il des hôpitaux où nous nous faisons soigner, des aides à domicile qui prennent soin de nos parents, des supermarchés où nous faisons nos courses ? Rien de tout cela ne pourrait fonctionner ! Un Français sur cinq est d’origine étrangère, et le fils d’immigrés juifs polonais que je suis a été meurtri par ces propos, comme la majorité des Français l’ont été.

voulez vous dépendre aussi du Rassemblement national ? Parce que nous ne voulons pas que notre pays vive sous la tutelle de l’extrême droite et parce que nous sommes responsables, nous avons accepté de discuter avec vous. Nous attendons du Premier ministre qu’il soit clair sur l’aide médicale de l’État (AME) et qu’il abandonne toute référence à la submersion migratoire ! La parole est

La question migratoire est source de tensions qui mettent à l’épreuve toutes les sociétés occidentales, et notre société n’y échappe pas. La traiter par le côté passionnel, c’est le meilleur moyen de ne jamais y répondre ; j’ai entendu que telle était aussi votre conviction.

étant, si nous regardons les choses en face, nous serons en mesure de maîtriser et d’accueillir correctement ceux qui viennent dans notre pays, comme c’est notre devoir. La question à résoudre, c’est la panne de l’intégration. L’intégration a été la dynamique singulière de la société française. Oui, elle est vécue par des millions de personnes, et en particulier par tous ces Français dont les ancêtres viennent de pays voisins ou lointains. est la vie de celles et de ceux qui accompagnent nos enfants et nos aînés, qui travaillent dans nos restaurants, des médecins dans nos services d’urgence, des informaticiens, des entrepreneurs – tous participent à la vie de notre pays et contribuent à sa richesse. Elle est aussi la vie de leurs enfants, qui vont à l’école. Les instruments d’une intégration réussie, nous les connaissons : le travail, la langue, les principes de la République, le principe de laïcité, c’est à dire notre héritage commun, humaniste – ce que nous devons transmettre. Mais tous ces instruments qui font notre fierté sont aussi pris dans la tourmente. Si nous améliorons notre éducation, si nous sommes fiers de nos principes, si nous sommes plus rigoureux et efficaces pour faire respecter la loi, alors l’intégration pourra être réussie.

Madame la ministre, à la fin de 2024, le chômage a connu sa plus forte hausse depuis dix ans, hors de la crise du covid 19 : +3,9 % par rapport au trimestre précédent ! Les jeunes de moins de 25 ans sont, malheureusement, les plus touchés. Ce chiffre est à mettre en regard du nombre record de défaillances d’entreprises. Toutes catégories confondues, ce sont plus de 6,2 millions de personnes qui étaient déjà enregistrées à France Travail il y a un an ! Derrière Derrière les statistiques, il y a autant de familles et de personnes seules, meurtries, qui aspirent à trouver un emploi et à vivre avec un salaire décent. Entendez vous les témoignages de ces salariés qui ont appris brutalement que la porte de leur entreprise était désormais fermée Beaucoup racontent qu’ils se sentent invisibles, mis de côté, bafoués. Et ce n’est pas fini ! Les indicateurs montrent que la situation va s’aggraver, une multiplication des plans sociaux étant 300 000 emplois pourraient être détruits prochainement. Cette situation catastrophique est la conséquence directe de la politique ultralibérale menée ces dernières années, et dont vous ne vous éloignez pas

La parole est à M. Georges Naturel, pour le groupe Les Républicains.

Cette ingérence intolérable, orchestrée par un régime totalitaire et ultranationaliste, classé parmi les plus corrompus au monde, constitue une tentative flagrante de déstabilisation de notre République et une atteinte inacceptable à notre intégrité nationale. Je regrette que les indépendantistes kanaks radicaux se discréditent en tombant dans le piège qui leur est tendu par des agitateurs à la solde d’une dictature hostile à la France et à ses valeurs de liberté. L’émancipation ne peut être revendiquée en s’alignant sur les initiatives d’une dictature et en cheminant à ses côtés ! Monsieur le ministre, il est impératif que la France, qui détient un siège au Conseil de sécurité des Nations unies, réagisse avec la plus grande fermeté, à la hauteur de l’affront qu’elle a subi. Quelles sanctions énergiques le Gouvernement entend il prendre contre l’Azerbaïdjan pour répondre à cette situation inacceptable et prévenir toute future ingérence qui menacerait la paix en Nouvelle Calédonie et dans l’ensemble de nos outre mer ?

Monsieur le sénateur, vous interrogez le Gouvernement sur les agissements coupables et intolérables du Baku Initiative Group, qui est installé en Azerbaïdjan et lié aux autorités Par des manœuvres numériques aussi bien que physiques, inauthentiques et malveillantes, qui visent nos régions, nos départements, nos collectivités d’outre mer, et en particulier la Nouvelle Calédonie, ce groupe a démontré sa volonté manifeste de s’ingérer dans notre débat public et de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, en l’occurrence notre intégrité territoriale et notre sécurité publique.

alors même que ses conditions de détention ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de Cécile Kohler et Jacques Paris, et alors même qu’il prenait le risque, en dénonçant ces conditions, de les voir se dégrader plus encore. Nous avons adressé des messages très fermes aux autorités iraniennes, leur expliquant

lundi dernier, à Bruxelles, lors du conseil Affaires étrangères, j’ai réclamé que l’Union européenne prenne des sanctions visant les responsables de ces détentions arbitraires. Notre mobilisation collective ne devra pas s’arrêter à la libération de ces trois otages. Il faudra également les accompagner par la suite.

adoption récente d’une loi pour obliger la France à décontaminer le Sahara des déchets nucléaires ; convocation de l’ambassadeur de France à Alger pour dénoncer de soi disant « traitements dégradants » d’Algériens à leur arrivée à Roissy ; remise en cause de notre ministre de l’intérieur et campagne de haine à son égard véritable prise en otage de l’écrivain Boualem Sansal, pourtant malade – et probablement très malade –, victime collatérale d’une relation bilatérale tendue, récemment retourné en prison après sa sortie d’hôpital et dont le seul délit est de se battre pour la liberté d’expression prise de position inimaginable, voire impensable, du recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui a osé se prononcer contre la résolution du Parlement européen du 23 janvier condamnant la détention de Boualem Sansal et réclamant sa libération immédiate et inconditionnelle.

comme le souhaite l’immense majorité des Français,

pour le groupe Union Centriste. Ma question s’adresse à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Combien de temps encore allons nous tolérer que les géants du numérique américains ou chinois défient ouvertement nos lois, mettent en danger nos enfants, manipulent les opinions et s’ingèrent dans nos processus électoraux pour saper nos démocraties ? L’activisme politique dangereux du propriétaire de X et le chantage inadmissible exercé par le président des États Unis sur la Commission européenne pour qu’elle abandonne enquêtes et sanctions vis à vis des plateformes appellent à des actions fermes et immédiates. Merci au Premier ministre espagnol Pedro Sánchez qui, à Davos, a appelé à « se rebeller » et à proposer des alternatives ! Pouvez vous nous dire, monsieur le ministre, quelle position et quelle stratégie la France entend défendre au sein du Conseil européen

avez évoqués. Plus que jamais, il est essentiel que la Commission européenne puisse faire respecter ces règles. Il y a quelques semaines, en Roumanie, l’élection présidentielle a dû être annulée parce qu’elle avait été perturbée

se livrent Américains et Chinois à coups de chiffres. Le programme cadre Horizon 2030 est défaillant ; il doit être rapidement révisé. Il lui manque un financement européen stratégique associant recherche et développement dans une logique, ainsi qu’une doctrine assumée de la commande publique visant à renforcer notre souveraineté. Il faut aussi rappeler à Mme von der Leyen que nos données sont un actif stratégique

du Congo (RDC) ne cesse de préoccuper la communauté internationale, sans pour autant que celle ci prenne une position claire, sans ambiguïté. À chaque action des milices, à chaque drame,

notre ambassade et plusieurs autres ont été les cibles d’attaques inadmissibles. Ces actes condamnables en disent long sur la perception par l’opinion locale de l’inaction de la communauté internationale face aux crimes de guerre commis en République démocratique du Congo.

viens aux événements survenus dans l’est de la République démocratique du Congo : la France condamne fermement l’offensive menée par le M23 et soutenue par les forces armées rwandaises,

et la politique de sécurité a à son tour condamné cette offensive et appelé à un cessez le feu immédiat. Vous le savez, jusqu’à présent, c’est le processus de Luanda qui a organisé la relation entre la RDC et le Rwanda, et c’est le processus de Nairobi qui a organisé la relation entre la RDC et les groupes rebelles, dont le M23. Ces médiations auraient dû porter des fruits, et il faut continuer de les soutenir. En tout état de cause, c’est par le dialogue et par la diplomatie qu’une solution sera trouvée

car à contretemps d’évolutions démographiques reconnues par tous. On est bien loin des engagements présidentiels de ne pas fermer de classe sans l’avis du maire. On est loin également des engagements des nombreux ministres de l’éducation nationale de construire des cartes scolaires pluriannuelles pour mettre fin à la gestion au jour le jour. Ces décisions prises dans l’opacité, à contre courant des engagements du Premier ministre, entretiennent la confusion et alimentent le désarroi des enseignants, des parents et des élus. À Paris comme dans le Lot, le Gers, la Somme, la Nièvre, le Nord, la Gironde, la Moselle – la liste est longue –, c’est l’incompréhension qui prévaut. Madame la ministre, ne laissez pas le désordre s’installer quand l’école a besoin, au contraire, d’un cap et de stabilité.

Je vous remercie de votre question, qui permet de clarifier quelques enjeux absolument essentiels. Ah ! Vous le savez, les moyens pour la rentrée 2025 ont été fortement revus à la hausse par rapport au projet de loi de finances déposé en octobre 2024.

avons nous proposé de maintenir les moyens de la rentrée dernière et de revenir intégralement sur les réductions de postes initialement prévues. Tel est notre objectif, et nous espérons que les conclusions de la commission mixte paritaire iront bien en ce sens. Comme vous, nous pensons que la baisse démographique doit être un levier pour améliorer l’école et pour réduire les inégalités, tant entre élèves qu’entre territoires ; tel sera le cas. Concrètement, à la rentrée 2025, les conditions d’apprentissage seront améliorées. Le nombre moyen d’élèves par classe, c’est à dire le taux d’encadrement, atteindra un niveau historiquement bas, inégalé depuis que cet indicateur est mesuré

Ce vote a été acquis avec l’avis favorable du gouvernement de Michel Barnier. Très bien ! Ma question est très simple : le gouvernement de François Bayrou est il du même avis, sur la même ligne ? Si oui, monsieur le ministre, quel est votre calendrier ? Il y a vraiment urgence

! Je vous répondrai donc très précisément. Quel calendrier ? Comme je l’ai indiqué tout à l’heure au sénateur Jean Yves Roux, je suis favorable à la différenciation territoriale, donc à la fin de l’obligation de transfert des compétences eau et assainissement des communes vers les EPCI. C’est clair !

d’autres, de graves dysfonctionnements cognitifs, des troubles cardiovasculaires, de l’épuisement, des dysfonctionnements musculaires, des anomalies immunologiques, des inflammations diffuses. La loi du 24 janvier

En janvier 2025, on nous annonce que les centres « covid long » n’ont plus de financement. Dans le Grand Est, quatre centres risquent d’être supprimés, les patients étant condamnés à l’errance médicale. Monsieur le ministre, que pouvez vous nous dire à propos de ces financements ?

médecin traitant peut trouver le centre de référence de proximité, au niveau départemental ou au niveau régional, où adresser les patients. Il a donc été institué une prise en charge

La séance est suspendue.

en prolongeant la jurisprudence de la Cour de cassation, qui admet que ces rôles ne conduisent pas nécessairement à provoquer la commission de l’infraction. Cet

permettra de renforcer les capacités d’enquête des forces de l’ordre, maillon essentiel des poursuites et des condamnations des auteurs d’infraction.

; les policiers infiltrés, qui font leur travail et qui sont tenus par la déontologie et les engagements qui sont les leurs ; les repentis qui vont sortir de la criminalité

L’État de droit impose aussi de s’assurer que les procédures respectant les droits de la défense soient prises en compte. Face à l’action publique, le mis en cause a des droits. Nous restons dubitatifs quant au sacrifice des droits de la défense afin de combler le manque de moyens de la justice pour faire son travail dans de bonnes conditions.

Le présent amendement vise à s’opposer à la réforme du régime des nullités prévue à l’article 20, qui restreint drastiquement le droit des parties à soulever des nullités de procédure. Le groupe GEST rappelle que les droits de la défense ont une valeur constitutionnelle. Le droit de soulever des nullités de procédure s’inscrit pleinement et légitimement dans l’exercice de ce droit fondamental. Ce droit est par ailleurs indispensable et vise à protéger les justiciables de décisions arbitraires. Le syndicat des avocats de France ajoute à ce sujet que le régime des nullités procédurales vient sanctionner le non respect de règles par les magistrats et les enquêteurs et constitue, de ce fait, une manifestation du principe d’égalité des armes, composante du droit à un procès équitable. La cause noble de la lutte contre le narcotrafic ne doit pas servir d’alibi pour déséquilibrer les droits des parties et le principe du contradictoire. Concentrer les efforts sur la lutte contre la propriété criminelle aura bien plus d’effets, à terme, sur le développement du narcotrafic que de s’attaquer aux droits de tous les justiciables.

sur le rapport de la commission d’enquête. Enfin, point qui fonctionne assez bien pour ceux qui connaissent ces matières en procédure civile et dont nous pensons qu’il peut aussi fonctionner en procédure pénale, lorsqu’une requête en nullité est faite, des mémoires sont échangés : le dernier mémoire doit récapituler l’ensemble des moyens de nullité, faute de quoi ils sont abandonnés.

qu’elle soit irrecevable.

aussi être analysé sous un angle constitutionnel : si nous décidons ici de choses aussi importantes que des simplifications de procédure pour, à la fin, se faire censurer par le Conseil constitutionnel parce que nous n’aurons pas respecté notre loi fondamentale, les services enquêteurs, les magistrats, la société auront été floués.

monsieur le ministre,

Cette clarification bienvenue permettra d’éviter des discussions sur ce qui est continu et sur ce qui ne l’est pas. Désormais, les choses seront limpides : le blanchiment est un délit continu et la poursuite n’intervient qu’à compter du jour où il est révélé.

Mme Isabelle Florennes. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est un outil utile pour préserver les juridictions de jugement d’une charge de travail parfois excessive. Elle permet

le champ d’application de ladite procédure, selon les conditions exigeantes prévues par le droit commun, à l’ensemble des crimes relatifs au trafic de stupéfiants, à l’exception de la direction et de l’organisation d’un réseau de trafic.

Narassiguin, sur l’article. Les auteurs de cette proposition de loi proposent, à l’article 21, de consacrer la compétence extraterritoriale des autorités françaises en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants. C’est évidemment Toutefois, je considère qu’il est tout aussi important, voire prioritaire de consacrer la compétence extraterritoriale en matière de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis à l’étranger.

Je m’adresse tout particulièrement à vous, monsieur le garde des sceaux : aujourd’hui, l’article 689 11 du code de procédure pénale comporte des verrous qui nous empêchent de juger les auteurs de tels crimes présents sur notre territoire, mais qui n’auraient pas de résidence habituelle en France.

à caractère personnel éventuellement révélées par les logiciels de rapprochement judiciaire à la clôture de l’enquête ou à l’expiration d’un délai de trois ans.

Le présent amendement vise à prolonger la durée de conservation des données jusqu’au terme de l’enquête, sous le contrôle d’un magistrat. Quel est l’avis de la commission ? Cette demande est à la fois utile et proportionnée

Le présent amendement vise un double objectif. En premier lieu, il tend à répondre à une asymétrie présente dans le code de procédure pénale, dont la rédaction actuelle n’autorise les perquisitions de nuit dans les locaux d’habitation en matière de criminalité organisée que dans le cadre de l’information judiciaire.

des garanties prévues en matière pénale et une limitation du dispositif aux seules infractions douanières graves et commises en bande organisée.

des perquisitions de nuit, dans des hypothèses bien définies – flagrance, risque de disparition des preuves –, avec une motivation renforcée. Dès lors que l’intervention du juge des libertés

Actuellement, la cosaisine des agents des douanes dans le cadre d’une enquête préliminaire aux côtés d’un service de police judiciaire est possible sous l’autorité d’un procureur de la République au motif que ces agents exercent une mission de police judiciaire. Mais ni le code des douanes ni le code de procédure pénale ne prévoient cette possibilité pour un juge d’instruction. Or la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a été confrontée à des situations procédurales dans lesquelles le concours de la douane n’a pu se poursuivre, alors que tel était le souhait partagé du service et de l’autorité judiciaire.

n° 76 rectifié. Cet amendement vise à permettre à des agents des douanes spécialement habilités de recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions. Si lesdits agents peuvent être cosaisis dans le cadre d’une enquête préliminaire, sous l’autorité du procureur de la République et aux côtés d’un service public judiciaire, une telle cosaisine est, en l’état du droit, exclue lorsque les investigations sont menées par un juge d’instruction, car ni le code des douanes ni le code de procédure pénale ne prévoient cette possibilité. Par cet amendement, nous proposons l’élargissement de la cosaisine des agents des douanes et des services de police judiciaire sous l’autorité d’un juge d’instruction, afin de conjuguer les compétences et la coopération entre les forces douanières et celles de la police judiciaire.

de vouloir réaffirmer que les agents des douanes peuvent être saisis ou cosaisis par le juge d’instruction dans le cadre des informations judiciaires. Nos auditions nous ont permis de constater qu’une telle possibilité, pourtant prévue par le code de procédure pénale, n’était pas effective faute de disposition miroir Les cosaisines fonctionnent parfaitement dans les enquêtes et ne soulèvent aucune difficulté, tant s’en faut. Il est donc judicieux que les juges d’instruction puissent, à l’instar des procureurs de la République, bénéficier de l’expertise des agents des douanes. C’est pourquoi

de corruption ou de menace liés à la criminalité organisée. Faire l’objet d’une enquête administrative est une procédure lourde, attentatoire à certaines libertés. Pour autant, et au regard de l’enjeu et de la dangerosité, ces travailleurs

Toutefois, puisqu’une telle enquête n’est justifiée que par le risque de corruption ou de menace lié à la criminalité organisée, l’enquête administrative doit y être explicitement cantonnée.

puissent faire l’objet d’un recours. Par souci de proportion, la personne bénéficiant d’une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation doit pouvoir exercer un recours contre la décision

prendre effet tant qu’il n’aura pas été statué en dernier ressort sur le litige. Le travailleur mis en cause ne peut être écarté que si le recours le confirme. Quel

Mme Audrey Linkenheld. Par cet amendement, nous souhaitons mieux protéger encore les personnes qui effectuent des signalements, notamment dans le cadre de la lutte contre la corruption,

Nous proposons donc de conserver les données de signalement sur un serveur sécurisé d’origine européenne, dont l’accès serait strictement réservé aux personnes habilitées, une procédure encadrée par décret,

des lanceurs d’alerte et efficacité de la lutte contre la corruption tout en assurant une sécurisation maximale des données sensibles.

dans le trafic de stupéfiants et, par extension, des compagnies qui les utilisent. La commission d’enquête a souligné dans ses travaux que les investigations menées sur des dossiers de trafic de stupéfiants par voie maritime avaient permis d’identifier des compagnies maritimes soit totalement factices, soit servant de façade à des organisations criminelles. Une telle mesure paraît donc nécessaire et bienvenue pour prévenir tout accès des narcotrafiquants aux ports français, qui constituent des infrastructures extrêmement sensibles et stratégiques dans la lutte contre le narcotrafic. l’avis de la commission ? Je suis très heureux de répondre à cette demande de notre collègue Pascal Martin, qui était membre de la commission d’enquête et qui nous accompagnait, notamment, sur les sites portuaires,

Cet amendement vise à compléter la palette de mesures prévues par l’article 22 pour lutter contre la corruption liée au narcotrafic dans les ports en permettant un recours renforcé à la vidéosurveillance, afin de détecter ces infractions.

s’appuyer sur la vidéosurveillance et d’en faire un outil précieux pour étayer des informations reçues ou pour lever le doute sur des faits liés au narcotrafic, par exemple des velléités de cession de badge nominatif à des fins crapuleuses, l’identification des véhicules venant déposer des individus à proximité des installations portuaires, des intrusions, qui nécessitent souvent une dépose près des ports, etc. Si le droit en vigueur n’empêche pas le préfet de demander la mise en place d’un système de vidéosurveillance au sein de l’installation portuaire, l’absence de définition d’un cadre juridique propre à ce dispositif constitue un vrai frein à son déploiement. Pour y remédier, le présent amendement vise à expliciter la possibilité pour le préfet de prévoir la conclusion d’une convention

Nous proposons que celles ci bénéficient des garanties suivantes : d’une part, une procédure contradictoire avant l’intervention de la décision en question ; d’autre part, l’obligation de motivation de ladite décision. Les nouvelles dispositions de cette proposition de loi relatives aux habitations et aux agréments des personnes physiques

– des personnels qui feraient l’objet d’un refus, d’un retrait ou d’une abrogation des agréments ou des habilitations pour accéder à une zone à accès restreint du port à la suite d’une enquête administrative de sécurité. La question des abrogations et retraits d’habilitation est déjà bien couverte par l’article 22 de la proposition de loi. Pour la mise en œuvre des enquêtes administratives de sécurité dans les ports, cet article renvoie aux conditions de droit commun prévues par l’article L. 114 1 du code de la sécurité intérieure, dont le III dispose précisément que ces décisions s’opèrent dans des conditions fixées aux articles L. 121 1 et L. 121 2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour les refus d’habilitation, le droit

Par cet amendement, élaboré à partir des réflexions de Transparency International France, nous souhaitons nous interroger sur le rôle des collectivités dans la prise en compte de la corruption.

La loi Sapin 2 décrit les mesures qui peuvent être prises en ce sens, comme les dispositifs de formation destinés aux cadres ou aux personnels, le dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements ou la cartographie des risques. risques. L’AFA, qui a été créée par la loi Sapin 2, est compétente pour contrôler la mise en œuvre d’un tel plan dans les entreprises et les administrations publiques. L’Agence, qui contrôle déjà les plus grandes collectivités, sans que les obligations de cette loi s’appliquent explicitement à celles ci, ci, recommande très fortement aux collectivités et aux administrations exposées au risque de corruption la mise en place de dispositifs de prévention. Tenant compte des constats et recommandations de l’AFA et des associations de lutte contre la corruption,

de cette nouvelle exigence, nous proposons d’instaurer des seuils pour les collectivités territoriales et de renvoyer à un décret pris en Conseil d’État le soin de définir le spectre des secteurs ciblés pour les administrations concernées.

loi permet déjà à l’AFA de contrôler les procédures mises en œuvre au sein des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des sociétés d’économie mixte. Le cas échéant, ces contrôles peuvent intervenir à la demande même de la collectivité. La systématisation de ce dispositif

tels que les services de sécurité intérieure, ou encore au sein des zones portuaires et aéroportuaires. Le rapport doit notamment étudier les causes endogènes des risques de corruption au sein de ces services. La commission d’enquête du Sénat a mis en lumière un phénomène grandissant et encore mal documenté de corruption des agents privés et publics. Il importe que l’État étudie avec sérieux les risques auxquels ces derniers sont exposés. Une telle étude ne serait pas complète si l’État ne prenait pas au sérieux les raisons qui expliquent la vulnérabilité de certains agents, notamment lorsqu’elles relèvent de sa propre responsabilité. Le niveau de Le niveau de rémunération de certains personnels publics ou les situations de sous effectif chronique de certains services, qui conduisent à une forme de désorganisation et à un défaut d’encadrement et de contrôle, sont des facteurs qui décuplent le risque de corruption. Le Parlement, déterminé à faire face à la menace de l’emprise du narcotrafic sur notre pays, doit être tenu informé de l’ensemble de ces risques et des facteurs de vulnérabilité auxquels sont exposés les services et les agents, afin de pouvoir effectuer un contrôle éclairé de l’action du Gouvernement et légiférer ainsi en toute connaissance

une évaluation de la gestion des téléphones portables en milieu carcéral et de l’efficacité des mesures prises pour limiter l’usage illégal de ces appareils. Je pense qu’il n’est point besoin

concernant la détention provisoire, la durée du mandat de dépôt et les règles en matière de demande de remise en liberté.

Toutefois, notre groupe n’est pas non plus favorable à l’allongement de la durée de la détention provisoire pour certains délits, qui n’est en fait justifié, comme l’a rappelé Jérémy Bacchi, que par l’engorgement des tribunaux Nous considérons qu’il n’est pas convenable de faire peser sur le justiciable les dysfonctionnements structurels de l’institution judiciaire. La procédure pénale et les principes qui l’irriguent ne doivent pas servir de variable d’ajustement pour pallier le manque de moyens matériels et financiers. Par ailleurs, une telle mesure n’aura sans doute que des effets marginaux, étant donné que le code de procédure pénale permet déjà de prolonger la détention provisoire en cas de trafic de stupéfiants, d’association de malfaiteurs, de proxénétisme, d’extorsion de fonds ou d’infraction commise en bande organisée, tandis que la durée maximale de la détention provisoire, à savoir deux ans, est inchangée.

M. Guy Benarroche. Cet amendement vise tout simplement à permettre la dématérialisation des demandes de remise en liberté, afin d’améliorer la fluidité de la procédure.

prévoyons la possibilité de faire usage de la visioconférence, même en cas de refus de la personne concernée, lorsqu’elle présente une dangerosité particulière. En ce qui concerne les demandes de mise en liberté,

Je crois que nous sommes d’accord sur ce point avec le Gouvernement. En outre, nous vous proposons de procéder également à trois aménagements procéduraux, qui ont donné lieu à beaucoup d’échanges. Nous souhaitons ainsi clarifier les dispositions relatives à la recevabilité des nouvelles demandes de mise en liberté, lorsqu’il n’a pas encore été statué

de répondre aux défis croissants liés à la sécurité carcérale, tout en garantissant un strict respect des libertés fondamentales. Ce dispositif, s’il était appliqué avec rigueur, pourrait constituer une avancée significative dans la lutte contre la criminalité en milieu pénitentiaire.

mais de fournir des outils ciblés, encadrés et proportionnés pour protéger les établissements pénitentiaires. Par cet amendement, nous souhaitons apporter une réponse pragmatique et équilibrée aux enjeux de sécurité carcérale, tout en respectant les exigences démocratiques et les libertés fondamentales.

une obligation de formation initiale pour les fonctionnaires pénitentiaires sur les risques de corruption et les moyens d’y répondre. La corruption en prison est un fléau sous estimé. Les établissements pénitentiaires sont particulièrement exposés aux tentatives de corruption, en raison de la proximité entre les détenus et les personnels, de la promiscuité des lieux et de la forte pression exercée par les réseaux criminels. Les formations ponctuelles, même si elles sont nécessaires, restent La formation initiale constitue un moment clé pour ancrer des réflexes professionnels et éthiques solides. Une meilleure préparation des personnels permettrait de réduire les vulnérabilités face aux pressions extérieures et d’améliorer la détection

Cette mesure s’inscrit dans la droite ligne de cette proposition de loi, qui vise à lutter partout contre le narcotrafic, et notamment dans les prisons, depuis lesquelles sont organisés nombre de trafics grâce à des téléphones pourtant interdits. L’adoption de cet amendement permettra de faciliter l’action des équipes pénitentiaires, dont je veux saluer le courage et le travail.

de l’information de l’administration pénitentiaire en cas d’installation d’une antenne relais à proximité d’un établissement pénitentiaire. Il s’agit d’un amendement de bon sens : on ne peut que s’étonner que l’administration pénitentiaire

graves, les réseaux de criminalité organisée ne reculant désormais devant aucun moyen pour permettre l’évasion d’une personne détenue au cours de son transport ou bien pour l’atteindre. Les agents de l’administration pénitentiaire de la prison de Perpignan – je sais, mes chers collègues, que vous avez les mêmes remontées partout sur le territoire national m’ont fait part de leurs craintes, pour ne pas dire de leurs peurs, lorsqu’ils doivent assurer ces convois. C’est dans cet esprit que j’ai déposé cet amendement qui a pour objet de doter l’administration pénitentiaire, à laquelle est désormais dévolue la responsabilité des missions d’extraction et de transfèrement, d’outils supplémentaires de surveillance et de protection. Ainsi, des caméras embarquées à bord des véhicules pourraient permettre de procéder à la captation d’images pendant les opérations de transport des personnes détenues, ce qui faciliterait le recueil de preuves aux fins de judiciarisation des incidents graves survenant sur la voie publique et la poursuite de de leurs auteurs. Mes chers collègues, en votant cet amendement, vous permettrez aux personnels de l’administration pénitentiaire, aux forces de l’ordre et aux magistrats de disposer d’un nouvel outil efficace et salutaire, à la fois dissuasif et répressif. Adopter un tel dispositif serait un signe fort dans la lutte contre le narcotrafic. Quel

Ces individus pris dans l’engrenage des réseaux criminels se retrouvent souvent sans perspective d’avenir, à la merci d’une exploitation quotidienne. Nous demandons au Gouvernement de remettre au Parlement dans dans un délai de six mois un rapport détaillant les solutions concrètes envisagées pour ces victimes. À l’heure où le plan social pour une réconciliation nationale n’est plus d’actualité, il s’agit de travailler sur des perspectives de sortie des réseaux, d’insertion sociale et professionnelle ou de rescolarisation. C’est un outil essentiel pour évaluer et ajuster nos politiques publiques. Nous ne pouvons ignorer les réalités sociales qui alimentent ces réseaux : précarité, déscolarisation, mal logement, dettes, rejet parental. Ce sont ces fractures que les trafiquants exploitent. Il est de notre devoir d’offrir à ces personnes un chemin vers la réinsertion et l’espoir d’une vie meilleure. J’y insiste, cette dimension sociale est aujourd’hui largement absente des politiques publiques de lutte contre la criminalité organisée. En mettant en lumière cette faille, nous espérons pousser l’État à pleinement assumer sa responsabilité envers les victimes des réseaux de narcotrafiquants, notamment les plus jeunes.

Je disais hier que j’avais la chance d’être invité partout dans le pays pour parler de ce sujet, comme Étienne Blanc, parce que beaucoup de maires sont très inquiets de ce qui se passe sur leur territoire.

non pas, si j’ai bien lu le texte, des trafiquants condamnés, mais des trafiquants suspectés. Il est déjà possible d’expulser de son logement social quelqu’un qui a été condamné

11 2 du code de la sécurité intérieure créé par l’article 24 de la proposition de loi. En effet, la peine d’emprisonnement de deux mois est insuffisante pour permettre au procureur de la République de traduire un contrevenant à une

troublent l’ordre public de manière grave ou répétée. Au regard de l’objet de la présente proposition de loi, et par souci de protection des locataires des HLM, il nous paraît indispensable de proportionner cette mesure. Ainsi, il est primordial qu’il soit explicitement précisé que les activités troublant l’ordre public de manière grave et répétée et qui justifient la résiliation du bail

privilégiée pour les narcotrafiquants. En effet, les habitations à loyer modéré peuvent servir de lieu de fabrication, de stockage et de vente de stupéfiants. L’illustration en a été faite dans ce débat.

Il devra porter un regard juste et critique sur la situation des HLM et ouvrir de véritables pistes de réflexion pour endiguer un phénomène majeur. Mes chers collègues, en votant cet amendement, vous offrirez aux bailleurs sociaux et aux élus locaux de nos territoires un début de réponse salutaire. Ces dérives inacceptables ne peuvent demeurer longtemps

! Cet avis est l’exception qui confirme la règle. Nous considérons que les bailleurs sociaux et le parc social locatif

Nous ne partageons pas le regard porté par le rapporteur sur cet amendement, dont nous souhaitons l’adoption.

Cet amendement vise à supprimer l’allongement de la durée de certaines techniques d’enquête, comme la géolocalisation et les interceptions téléphoniques. Parmi elles figurent notamment la durée maximale d’autorisation de ces techniques et le contrôle que peut exercer un juge. Enfin, l’amendement tend à supprimer la possibilité de régulariser la mise en place d’une géolocalisation par une décision intervenant dans un délai maximum de huit heures.

au principe du contradictoire et aux droits de la défense. L’atteinte aux droits de la défense réside dans le fait que, les parties n’ayant pas accès à ces informations, elles se trouvent dans l’impossibilité de formuler d’éventuelles critiques quant à la légalité de ces actes. Le Conseil constitutionnel s’est prononcé, dans une décision du 25 mars 2014 – citée à l’instant par le ministre d’État – sur une technique de procès verbal distinct similaire appliquée pour la géolocalisation. Les Sages ont jugé que cette technique était conforme, car les parties disposent d’un délai de dix jours pour demander au président de la chambre de l’instruction de contrôler le recours à la procédure. Un recours similaire existe aussi pour les témoignages anonymes. Or le dispositif proposé n’a pas intégré ce recours.

de l’interdiction de prononcer une condamnation sur le seul fondement des éléments de géolocalisation recueillis. Les juges ont ainsi considéré qu’une information mettant en cause une personne ne peut pas constituer un élément de preuve devant la juridiction répressive

requête. Cet amendement a pour objet de faciliter la possibilité pour nos enquêteurs d’entrer dans les systèmes de communication protégés des narcotrafiquants. Quel est l’avis de la commission ? Il est

l’amendement n° 25 rectifié. Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs spéciaux d’enquête que peuvent mobiliser les agents des douanes pour s’adapter aux nouveaux moyens de télécommunication des narcotrafiquants. pour objet d’octroyer aux agents des douanes habilités la possibilité de déclencher à distance la captation, la fixation et l’enregistrement de paroles prononcées ou d’images intégrées aux matériels numériques utilisés par un ou plusieurs mis en cause. La

les infractions. Il n’est pourtant que très marginalement mobilisé par l’autorité judiciaire pour lutter contre le blanchiment du produit des infractions à la législation sur les stupéfiants. amendement a pour objet de permettre aux parquets et aux juges d’instruction de confier plus aisément à l’Onaf les enquêtes portant sur ces infractions et de mobiliser son expertise sur le blanchiment lorsque les enquêtes sont diligentées à la suite d’une constatation réalisée par des agents des douanes. des douanes. Faciliter la saisine de l’Onaf en matière de blanchiment de trafic de stupéfiants, après une constatation réalisée par les agents des douanes, permet de supprimer dans la loi une distinction qui n’est plus adaptée à l’origine diverse des fonds blanchis par les organisations criminelles.